La séance est ouverte. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2018 ! Le compte rendu intégral de la séance du 20 décembre 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Guy Besse, qui fut sénateur de l'Indre de 1982 à 1989, et Georges Othily, qui fut sénateur de la Guyane de 1989 à 2008. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant les ordonnances du 3 août 2016, qui s'est réunie le mercredi 20 décembre 2017, est parvenue à l'adoption d'un texte commun. J'informe le Sénat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

de déménager son centre de recherche et de développement de Galderma, situé à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. Après trente-six ans de présence dans ce département, le plus grand centre de recherche du groupe devrait disparaître en septembre prochain. menacés. Si une centaine d'opportunités professionnelles sont proposées en Suisse à travers un plan de mobilité internationale, nombre de salariés risquent de perdre leur emploi en France. Certains ne pourront évidemment pas accepter la mobilité en Suisse, en raison de leur implantation locale dans les Alpes-Maritimes, où leurs conjoints travaillent et où leurs enfants sont scolarisés. Le plan actuellement négocié entre la direction et le comité d'entreprise n'apporte pas de réponse satisfaisante, s'agisse des indemnités, de la formation pour d'éventuelles reconversions ou de la prise en compte de l'ensemble des situations individuelles. Je pense en particulier aux salariés en situation de handicap et aux salariés dits « seniors », qui présentent malheureusement les taux d'embauche les plus faibles. Si Nestlé a annoncé être prêt à céder la propriété intellectuelle pour faciliter la création de start-up sur le site, ce changement de statut peut se réduire à un mirage : il n'offre pas les mêmes garanties professionnelles qu'une entreprise internationale, internationale, surtout pour des scientifiques. Enfin, la recherche d'un repreneur se révèle plus que nébuleuse. Seule l'arrivée d'une entreprise équivalente,

qui a exprimé toute l'attention de l'État aux salariés de Galderma. Mais, à ce jour, ces derniers n'ont toujours aucune visibilité au sujet d'éventuels repreneurs. Pourtant, depuis la loi dite « Florange » de 2014, les entreprises qui cessent leur activité ont des obligations de recherche de repreneur, d'information et de dialogue social. L'État a donc une responsabilité de suivi. Où en est-on, concrètement, dans la recherche d'un repreneur ? L'État a-t-il des propositions ?

la société Galderma, située à Biot, à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, oeuvre dans le domaine de la recherche et développement. Depuis 2016, elle est propriété à 100 % du groupe Nestlé. Le projet de réorganisation mondial lié à l'abandon des produits de type « crème » s'accompagne à terme du désengagement du groupe de son site de Sophia Antipolis, avec les conséquences et les inquiétudes que vous avez décrites. de sauvegarde de l'emploi, ou PSE. Dans un premier temps, un plan de départs volontaires porte sur 400 postes, l'entreprise proposant seulement 100 postes de reclassement au niveau de son siège, en Suisse. La première consultation du comité d'entreprise a eu lieu le 2 octobre

il a répété une fois encore combien le Gouvernement est attaché à la recherche d'un repreneur pour l'ensemble du site et au respect des dispositions de la loi Florange. Ce projet devra aboutir au repositionnement d'activités de pointe, qui sauront tirer parti des compétences de haut niveau dont disposent les salariés du site. les salariés du site. M. Floris poursuit ses discussions avec le groupe Nestlé. Il se rendra dans votre département le 7 février prochain pour faire le point sur les projets de reprise du site avec la direction et les représentants du personnel, que nous lui avons demandé de rencontrer.

à la mise en oeuvre de cette réorganisation, à la recherche d'activités nouvelles et aux mesures d'accompagnement qui seront proposées aux salariés. L'ensemble de ces démarches devront être à la hauteur des capacités d'un groupe comme Nestlé.

afin d'assurer un véritable maillage territorial et de soutenir l'économie locale. Ces collectivités territoriales, touchées par la baisse des dotations de l'État, sont confrontées au problème de l'importance de l'autofinancement pour faire aboutir leurs projets.

Si tel est le cas, seront-ils remplacés par de nouveaux accompagnements financiers tout aussi avantageux ? J'insiste encore, monsieur le secrétaire d'État, sur l'importance de ces dispositifs pour les collectivités, soucieuses de maintenir leurs investissements et, partant, l'attractivité de leur territoire. La parole

l'économie et des finances a récemment confirmé au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations la prolongation jusqu'en 2020 de l'enveloppe de 20 milliards d'euros en faveur du secteur public local. Une rationalisation des dispositifs publics de financement du secteur public local paraît toutefois nécessaire. la Cour des comptes a récemment appelé l'attention du Gouvernement sur la nécessité de rationaliser les dispositifs publics locaux de financement, dans un contexte de taux extrêmement favorables pour les collectivités territoriales et de concurrence entre plusieurs dispositifs,

être le dispositif public pivot de l'offre de prêt. Pour ces raisons, l'enveloppe est tarifée au taux du livret A assorti d'une marge de 130 points de base et recentrée sur les prêts de long terme, soit vingt-cinq ans et plus, pour lesquels la ressource du fonds d'épargne, qui n'intervient qu'à taux variable, contrairement aux autres dispositifs publics et aux banques commerciales, paraît compétitive dans la durée. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre du Grand plan d'investissement, le ministre a souhaité ouvrir, pour cinq ans, une enveloppe de 2 milliards d'euros à taux préférentiel, destinée au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics, conformément aux recommandations du rapport établi par M. Pisani-Ferry à la demande de M. le Premier ministre. Cette enveloppe, qui remplace l'actuelle enveloppe de prêts « croissance verte », sera tarifée au taux du livret A majoré de 75 points de base et pourra financer des projets d'une maturité minimale de vingt ans.

les communes ayant souscrit à l'époque un tel prêt à taux fixe consacrent tous les ans plusieurs dizaines de milliers d'euros, pris sur leur budget de fonctionnement, au paiement des intérêts de ce prêt.

contrairement aux banques ordinaires, la Société de financement local, la SFIL, qui a repris la gestion des prêts aux collectivités territoriales à la suite de la déconfiture de Dexia, s'en tient strictement aux clauses du contrat signé et réclame une indemnité de sortie anticipée véritablement léonine. Ainsi, pour la commune dont j'ai parlé, la SFIL exige plusieurs centaines de milliers d'euros, correspondant pratiquement à tous les intérêts restant à payer jusqu'à l'échéance du prêt. Cette situation est totalement inacceptable. Ces communes, déjà mises en difficulté par l'importance de leurs frais financiers, subissent de ce fait une double peine.

compte tenu de ces éléments, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer les mesures que pourrait prendre le Gouvernement pour permettre à ces collectivités territoriales de sortir d'une situation particulièrement néfaste

Compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt, les établissements de crédit sont aujourd'hui exposés à des pertes actuarielles potentiellement importantes, ce qui explique le niveau élevé des indemnités de remboursement anticipé qu'ils demandent souvent aux collectivités.

La renégociation éventuelle des contrats en cours demeure, en principe, du ressort des parties prenantes que sont l'établissement de crédit et la collectivité territoriale concernée, dans le respect de leurs intérêts mutuels. Nous appelons donc au dialogue entre les collectivités territoriales emprunteuses et les banques prêteuses ; mais, en l'état actuel des choses, l'État ne peut pas s'immiscer dans leurs relations contractuelles.

Tous les dépôts effectués sous forme papier sont désormais renvoyés aux déposants, sans enregistrement, ce qui constitue une violation du traité international sur le droit des marques signé le 27 octobre 1994 et ratifié par la France,

voire sur le plan international, à rejeter les formalités sur support papier. Or l'article 63 du règlement délégué 2017-1430 de la Commission du 18 mai 2017

autorise de tels dépôts. Le Défenseur des droits, dans son rapport du 30 mars 2016 sur l'accès aux droits, rappelle clairement les risques de fracture numérique à l'égard des services publics pratiquant la « tout-numérisation le secrétaire d'État, pouvez-vous m'indiquer si le Gouvernement a l'intention d'agir pour que la continuité du service public de cet établissement soit assurée par la réception, l'enregistrement et le traitement des dépôts sous forme papier de marques, dessins et modèles et d'inscriptions aux registres de la propriété industrielle ? La parole

L'objectif est de simplifier et de faciliter l'accès de nos concitoyens aux services publics en leur offrant un service plus rapide et plus efficace. L'Institut national de la propriété industrielle s'inscrit dans cette dynamique commune à tous les services publics. Grâce aux téléservices mis en place, le dépôt en ligne et la suppression des formalités au format papier sont effectifs pour les indications géographiques et les demandes d'extension des marques à l'international depuis 2015, pour les oppositions de marques depuis 2016 et pour les marques, les dessins et modèles et les inscriptions modificatives depuis octobre 2017. La dématérialisation complète de ces procédures présente de nombreux avantages. Ainsi, l'utilisation du support électronique rend plus fluide le traitement des dossiers, ce qui bénéficie en retour au déposant, lequel peut obtenir une réponse plus rapide à sa demande. Les téléservices renforcent la qualité des échanges entre l'INPI et les déposants, en permettant notamment à ceux-ci d'avoir accès en temps réel à l'état d'avancement de leurs demandes. Enfin, le dépôt électronique élimine le risque d'erreur de saisie des données et sécurise ainsi la procédure de traitement des dossiers. Des mesures d'accompagnement ont été prises pour faciliter l'appropriation des téléservices par les utilisateurs. Ainsi, l'institut propose à tous les déposants une assistance téléphonique personnalisée par des spécialistes pour les aider dans leur prise en main. Les équipes des délégations régionales de l'INPI, implantées dans chacune des treize régions métropolitaines, sont également disponibles pour proposer leurs services et fournir tous les renseignements utiles. L'INPI reçoit annuellement plus de 90 000 demandes de marques françaises, dont 94 % étaient déjà déposées sous un format électronique avant le mois trois mois après la décision de dématérialisation complète de la procédure, l'INPI reçoit moins d'un dossier par jour par voie papier sur les 400 marques déposées quotidiennement, soit 0,25 %, ce qui permet d'apporter aux usagers dans cette situation une réponse personnalisée.

Envisagez-vous de procéder à une étude approfondie de ces différentes situations, afin d'en évaluer la portée et les conséquences ? Plus encore, comptez-vous engager une réflexion afin d'annuler ces amputations sur les budgets des communes qui ne perçoivent aucune DGF et qui doivent faire face à de nouvelles baisses de recettes, notamment lorsqu'elles

Depuis 2014, une contribution au redressement des finances publiques, ou CRFP, a ainsi été répartie entre les différentes catégories de collectivités, et ce proportionnellement à la part respective de leurs recettes dans les recettes totales des collectivités

simplement en cas d'insuffisance de la dotation forfaitaire que les communes ont contribué au redressement des finances publiques un prélèvement sur recettes fiscales. Cette situation concernait 439 communes au total en 2017. Le prélèvement sur la fiscalité ne pouvait donc concerner que des communes pour lesquelles la dotation forfaitaire représente une part faible des ressources. C'est le cas de la commune de Gandrange que vous avez citée en exemple, pour laquelle la dotation forfaitaire représentait seulement 5 % des recettes en 2014. Sur le fond, le choix d'un vecteur complémentaire d'imputation de la CRFP a été fait par le législateur dans le souci de garantir l'égalité entre les collectivités.

C'est également la raison pour laquelle le législateur a fait le choix, à travers l'article 159 de la loi de finances initiale pour 2018, de reconduire à compter de 2018 les prélèvements opérés sur la fiscalité des communes au titre de la CRFP, comme cela était prévu depuis 2014. Là encore, annuler ces prélèvements après 2017 aurait conduit les communes ayant payé une partie de la contribution sur leurs recettes fiscales à bénéficier d'un avantage sous la forme d'une sorte de « remise à zéro » des compteurs, alors que la contribution a été intégrée dans la base de calcul de la DGF au second point de votre question. Les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des concours financiers et des fonds de péréquation prennent bien en compte le rétrécissement des bases fiscales lié à d'éventuelles restructurations d'entreprises.

le 15 octobre 1985 par le Conseil de l'Europe. Ne pensez-vous pas que la décision d'amputer les ressources propres des collectivités locales, afin d'abonder le budget de l'État et de diminuer son déficit, obère la capacité de ces collectivités à

part, notre législation et, de l'autre, le droit européen applicable, notamment l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale, en vertu duquel « les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement

des centres experts innovants qui travaillent sur la schizophrénie, les troubles bipolaires ou encore le syndrome d'Asperger, un centre de remédiation cognitive et sociale et un service d'addictologie. D'une capacité de cent lits, le pôle psychiatrique a enregistré 41 41 000 journées d'hospitalisation en 2017 et se trouve aujourd'hui au bord de l'explosion : unités suroccupées, manque de lits, sous-effectif du personnel,

Je pense notamment à l'hôpital psychiatrique de Rennes ou au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon, dont on connaît les mobilisations. L'équipe de direction de l'hôpital Albert-Chenevier a tiré la sonnette d'alarme quant à la dégradation des conditions de travail des soignants et de la prise en charge des patients, lesquels demandent peut-être encore plus que d'autres de l'attention, de la bienveillance, du temps d'écoute et un cadre serein.

l'hôpital Chenevier héberge trois secteurs de psychiatrie : Maisons-Alfort, Créteil et Bonneuil-Boissy-Saint-Léger. Ces secteurs interagissent avec trois groupements hospitaliers de territoire : le GHT 94 Nord, le GHT 94 Est et le GHT 94 Ouest.

un service d'accueil des urgences psychiatriques, qui recense 3 300 passages par an et dessert la quasi-totalité des urgences psychiatriques du Val-de-Marne. Un tiers des passages concerne les secteurs de l'hôpital Chenevier, deux tiers d'entre eux concernent le Val-de-Marne.

de l'hôpital Henri-Mondor, dont la mission est de prendre en charge les soins intriqués, somatiques et psychiatriques, ainsi que les primo-suicidants. Ce nombre de lits est structurellement faible et le taux, assez bas dès l'origine, est pénalisé par l'accroissement de la population desservie. Le taux d'occupation est de 95 % ; la durée moyenne de séjour est bonne, mais s'allonge ; le taux des hospitalisations sous contrainte a été multiplié par deux en cinq ans, et le taux de réhospitalisation est de près de 22 %. La réponse à cette tension dont l'hospitalisation complète fait l'objet se trouve en partie dans le déploiement de structures extra-hospitalières. médico-psychologiques, ou CMP, installés à Créteil et à Boissy-Saint-Léger, et d'un dispositif de soins partagés destiné à faciliter le lien avec les médecins généralistes et les spécialistes de ville.

Les moyens humains notifiés au pôle de psychiatrie ont été substantiellement accrus en 2016 pour faire face à ces missions. Nous souhaitons qu'ils soient maintenus. Cependant, on note une réelle difficulté dans les recrutements d'infirmiers. Cette situation est née d'un contexte général de recrutements en tension. Le problème est encore

sur la situation sanitaire très préoccupante que connaît le département du Pas-de-Calais. Ainsi, sur le plan de la démographie médicale, on note une diminution du nombre de médecins généralistes libéraux et une augmentation significative de leur moyenne d'âge, ce qui entraînera inéluctablement un important mouvement de départs à la retraite dans les prochaines années. À titre d'illustration, les agglomérations de Lens-Liévin et de Béthune-Bruay apparaissent moins dotées en médecins généralistes et spécialistes que d'autres agglomérations de même importance. À terme, il existe clairement un risque de désertification médicale. Le taux d'équipement de santé du territoire à l'échelle du pôle métropolitain de l'Artois, par exemple, montre un sous-équipement en centres de médecine préventive et en établissements de court et moyen séjours. La situation des hôpitaux dans le Pas-de-Calais est très préoccupante les services des urgences sont saturés et les personnels sont à bout de forces. Au-delà de ces difficultés conjoncturelles, c'est la situation du centre hospitalier de Lens à l'horizon 2020 qui inquiète les personnels, du fait de la diminution annoncée du nombre de lits. La disparition du service de pneumologie de cet hôpital est une nouvelle illustration de la crise sanitaire qui affecte le Pas-de-Calais. L'inquiétude est très forte chez les patients concernés par cette fermeture, d'autant qu'ils se retrouvent parfois sans suivi, sans prise en charge, alors même que, dans le département, le nombre d'affections pulmonaires est bien supérieur à la moyenne nationale. En outre, les menaces pesant sur le service de cardiologie de l'hôpital de Béthune amplifient l'impression ressentie par la population d'être sacrifiée sur l'autel des économies budgétaires dans le domaine de la santé.

dans le domaine de la santé. Quelles mesures concrètes entend-il mettre en oeuvre pour répondre à l'urgence sanitaire affectant le département du Pas-de-Calais ? Dans un souci d'optimisation, une mutualisation pourrait être envisagée, qui s'appuierait sur le futur centre hospitalier de Lens, dit « hôpital numérique pilote ». Ainsi, un regroupement multipolaire Lens-Béthune-Arras-Douai permettrait d'élargir cette excellence, de voir revenir nos médecins et d'assurer le service qu'attendent nos concitoyens ! La parole

Le développement de l'attractivité constitue donc l'un des principaux enjeux de ce territoire pour les cinq prochaines années. Il s'agit pour nous d'accompagner les professionnels de santé tout au long de leur parcours et de les attirer dans les territoires et les disciplines les plus en tension. Quatre priorités ont été identifiées dans le Pas-de-Calais accompagner l'installation des professionnels de premier recours et soutenir les dynamiques de regroupements pluriprofessionnels et de télémédecine, afin de lutter contre l'accentuation des inégalités infra-territoriales- à ce titre, une attention particulière est portée aux zones rurales du Montreuillois, du Ternois, du sud-Arrageois et du sud-Audomarois ; ensuite, diminuer le recours aux services d'urgence en développant les maisons médicales de garde et en communiquant sur la bonne utilisation du système de soins ; en outre, conforter l'offre de formation paramédicale et médicale de proximité ; enfin, améliorer l'attractivité du Pas-de-Calais pour les psychiatres et les pédopsychiatres.

Lors du conseil de surveillance du 17 octobre 2017, la fermeture du service de pneumologie, qui regroupe 15 lits, a été annoncée à compter du 1 novembre 2017. À cette date, il ne restait que deux pneumologues dans l'établissement. Dans un premier temps, et pour remédier à l'urgence, des décisions ont été prises afin d'assurer la continuité des soins au centre hospitalier de Lens avec une astreinte de pneumologie vingt-quatre En parallèle, et pour apporter une réponse à long terme, l'agence régionale de santé, l'ARS, accompagne les pneumologues de Lens et de Béthune pour mettre en place une organisation territoriale de la pneumologie. Un travail comparable est également en cours pour la cardiologie. Dans la perspective de la constitution de ces deux équipes médicales de territoire, l'ARS a décidé d'allouer un financement exceptionnel de 500 000 euros. J'ajoute que l'amélioration de l'attractivité de ce territoire pour les professionnels passe par une dynamique partenariale plus forte entre les acteurs au sein des GHT, sans exclure la poursuite des coopérations préexistantes avec les autres partenaires. Les travaux conduits pour l'élaboration des projets médicaux partagés des GHT dans le territoire du Pas-de-Calais témoignent d'ailleurs d'une volonté de travail en commun qui répond à cette exigence et que le Gouvernement souhaite accompagner.

Ma question porte sur la nécessité pour le législateur, les agriculteurs et les citoyens de pouvoir connaître la dangerosité du glyphosate et, surtout, d'assurer la traçabilité de ce produit. En effet, face à des études scientifiques contradictoires, il faut appliquer le principe de précaution, comme le Président de la République s'y est engagé. La mise en oeuvre de ce principe réduit néanmoins la compétitivité de notre agriculture et n'atteint pas le but visé, à savoir la protection de la santé des consommateurs, si des produits importés contenant du glyphosate restent disponibles. Dans ce cas, les consommateurs français, de même que nos agriculteurs, qui se verraient interdire l'usage du glyphosate sans solution équivalente, seraient floués.

Par ailleurs, l'utilisation massive du glyphosate a des conséquences sur le plan environnemental : on constate la présence de cette substance dans les cours d'eau et dans ses produits de décomposition. C'est dans ce contexte que le gouvernement français s'est opposé à l'approbation longue proposée par la Commission européenne. Le Gouvernement a souhaité que la durée de réapprobation soit strictement limitée à celle qu'exigent la recherche, l'identification et la diffusion de pratiques alternatives. À cette fin, il a été demandé à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, de produire un rapport sur les usages du glyphosate et sur ses alternatives. Le rapport remis par l'INRA le 1décembre 2017 montre que des solutions de substitution existent pour certains usages du glyphosate, mais qu'un important travail de recherche et de diffusion d'alternatives est nécessaire pour d'autres usages.

Les efforts déployés pour le changement des pratiques agricoles doivent être récompensés et valorisés par une meilleure structuration de l'aval et une plus grande information des consommateurs. Des contrôles très réguliers des services de l'État, notamment de la direction générale

L'orientation doit s'entendre tout au long de la vie. Chaque individu est appelé à effectuer plusieurs choix au cours de son parcours scolaire et professionnel. Or, entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, il y a comme qui dirait un trou dans la raquette À partir de trente ans, point de reconversion possible ; certes, les formations existent, mais les recruteurs restent bloqués par l'existence des charges afférentes. Pour plus d'efficacité, il faudrait selon moi créer un statut unique de l'apprentissage en France. Aujourd'hui, il existe des centaines d'accords de branche ; le coût horaire n'est jamais le même, la prise en charge non plus. explique aussi la désaffection des chefs d'entreprise pour l'alternance. Il faudrait également exonérer de toutes les charges patronales et fixer les salaires uniquement en fonction de l'âge. Actuellement, les salaires sont fixés à la fois en fonction de l'âge et de la branche. Auparavant, le salaire des apprentis était calculé sur la base désormais, il l'est en fonction des conventions de chaque branche, ce qui a considérablement augmenté le coût pour les entreprises. Développer l'apprentissage nécessite un engagement collectif de l'État, des régions, des partenaires sociaux et des autres acteurs concernés, dans un contexte où la taxe d'apprentissage, qui finance d'autres formations initiales,

Vous le savez, les deux contrats de travail en alternance que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation ne répondent pas aux mêmes besoins et ne visent pas les mêmes buts. En effet, le contrat d'apprentissage répond aux besoins de formation initiale et a pour but l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, alors que le contrat de professionnalisation, qui relève de la formation continue, participe à l'insertion ou à la réinsertion dans l'emploi. Nous constatons aussi des différences notables dans la mise en oeuvre de ces deux contrats. Ainsi, la durée du contrat de professionnalisation est stable et s'établit aujourd'hui à 13,7 mois, alors que le contrat d'apprentissage est de 20 mois. Les secteurs d'activité sollicitant ces deux contrats diffèrent eux aussi sensiblement. Les secteurs de la banque, des établissements financiers et d'assurances, le commerce, les bureaux d'études et prestations de services aux entreprises et le secteur sanitaire et social font plus appel, en part relative, aux contrats de professionnalisation. Il convient néanmoins de noter que le plafond d'âge d'éligibilité à ces contrats a été fortement relevé, Ils permettent donc la prise en charge de nombreuses personnes. En effet, au-delà de l'expérimentation d'entrée en apprentissage jusqu'à trente ans lancée le 1 janvier 2017, il existe des dérogations légales permettant des reconversions plus tardives dans certains domaines. Ainsi, il est possible de signer des contrats d'apprentissage indépendamment de la limite supérieure d'âge pour les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, pour les personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise, si le projet est subordonné à l'obtention d'un diplôme, ou encore pour les personnes bénéficiant d'un statut de sportif de haut niveau.

même si, à ce jour, fort peu de conventions collectives prévoient des grilles particulières. Seuls les apprentis de plus de vingt et un ans sont actuellement soumis à une base de calcul d'un éventuel salaire de base conventionnel.

La rémunération de l'apprenti, les modalités de gestion du contrat d'apprentissage et une meilleure complémentarité des deux contrats en alternance sont abordées dans le cadre de la concertation, afin que l'alternance puisse bénéficier à tous dans des conditions optimales. Nous sommes tous persuadés que l'alternance et l'apprentissage font partie des

à vingt-cinq ans lors de la journée défense et citoyenneté. Ils sont inacceptables dans une société où l'instruction est obligatoire. Il apparaît, constat identique depuis plusieurs années, que, plus les indices de pauvreté sont bas, plus celui de l'éducation est faible. on avait annoncé « des efforts importants entrepris, traduits dans le programme de travail pour la période 2014-2017 », comprenant notamment « des actions de formation d'envergure à destination des enseignants et des actions spécifiques à l'intention des jeunes ». Le décalage dont souffre la Picardie, et plus particulièrement l'Aisne, par rapport à la situation nationale ne s'est pas estompé en l'espace de quinze

politiques publiques éducatives, rapport au titre troublant : Dernière ces chiffres, ces pourcentages ou ces statistiques, nous parlons de nos concitoyens, qui seront de moins en moins armés pour affronter les difficultés en vue de trouver une formation ou un travail et d'assumer dignement l'entretien d'une famille. N'est-il pas temps de nous inspirer de nos voisins du nord de l'Europe, de l'Allemagne, voire de la Corée,

de dédoubler les classes primaires dans les zones défavorisées, et nous vous en louons. J'ai bien entendu votre réponse lors de l'examen du budget 2018, pour ce qui concerne la détection et la prévention des élèves atteints de troubles « dys » par une médecine scolaire

En parallèle, plusieurs mobilisations sont prévues, dont certaines étaient mentionnées dans votre question. L'école maternelle va faire l'objet d'une réflexion et de transformations, afin qu'elle soit, plus encore qu'aujourd'hui, l'école de l'épanouissement et de l'apprentissage du langage. Vous le savez, au mois de mars prochain auront lieu des assises de la maternelle, qui seront présidées par Boris Cyrulnik. Ces dernières vont nous permettre de prendre, dès la rentrée prochaine, un certain nombre de mesures en faveur de l'école maternelle.

renforcées, en partenariat avec les communes concernées. Vous le savez, l'académie d'Amiens est particulièrement mobilisée sur ces questions. Je m'y suis déjà rendu à plusieurs reprises depuis ma prise de fonctions, avec une priorité clairement affichée, à savoir l'acquisition des savoirs fondamentaux

Monsieur le ministre, la décision du Gouvernement de supprimer un nombre très significatif de contrats aidés, près de 40 % par rapport à l'année 2016, suscite de vives inquiétudes dans de nombreuses associations, particulièrement dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire.

la diminution des dotations aux collectivités territoriales, la suppression de la taxe d'habitation, qui ne permettra plus aux communes de développer une fiscalité propre sur leur territoire, enfin la suppression de la réserve parlementaire, dont 70 % des fonds venaient soutenir des projets associatifs dans les territoires, toutes ces mesures frappent en premier lieu, et directement, les structures associatives.

pose de véritables problèmes de garde pour les parents, particulièrement dans les familles les plus modestes. Or, le secteur associatif, c'est 1,3 million d'associations, 13 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés qui structurent en profondeur notre pays représente 85 milliards d'euros de budget, soit 3,5 % de notre PIB. On le constate, les associations sont une richesse pour la Nation. Il ne s'agit donc pas d'opposer emploi aidé et emploi qualifié et de ne retenir que le caractère économique pour juger de l'efficacité de ce dispositif. Le tissu associatif est en effet indispensable dans les quartiers pour maintenir le lien social, favoriser le vivre-ensemble et le dialogue civil. Aussi, alors que, pour la première fois depuis 1957, un ministère de plein exercice ne fait plus référence à la jeunesse et à la vie associative, je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir prendre en compte la spécificité du secteur de l'accueil de notre jeunesse. La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale.

mais elle ne pouvait être différente pour un gouvernement qui veut changer les mauvaises habitudes consistant à construire des budgets non sincères en début d'année, qu'il faut revoir à mi-parcours et qui, de surcroît, ne permettent pas de conduire des politiques que vous et vos collègues parlementaires votez.

Le Gouvernement en est tout à fait conscient. C'est pourquoi nous avons revu le volume des contrats aidés à la hausse par rapport à la loi de finances initiale pour 2017, en dépit du contexte de contrainte budgétaire. 280 000 contrats aidés avaient été programmés pour l'année, mais les deux tiers de cette enveloppe annuelle ont été consommés dès le premier semestre. Il faut sans cesse le rappeler, face à un certain nombre de discours Le Gouvernement a accordé une rallonge dans le contexte de maîtrise du déficit. Il a ainsi souhaité porter cette enveloppe à 320 000 contrats aidés sur l'année, soit 40 000 emplois de plus que ce qui avait été prévu. Par ailleurs, de manière opérationnelle, cet effort a conduit le Gouvernement à cibler quatre secteurs prioritaires pour la fin d'année 2017 : l'éducation nationale et plus particulièrement l'accompagnement des élèves en situation de handicap ; l'outre-mer ; l'urgence sanitaire et l'urgence sociale, c'est-à-dire le secours alimentaire et l'hébergement social. Pour le secteur associatif, les contrats aidés ont donc été concentrés sur l'urgence sanitaire et sur l'urgence sociale, notamment parce qu'en période hivernale l'aide alimentaire, l'accompagnement social ou l'hébergement, en particulier médicalisé, des personnes dépendantes, sans abri ou atteintes d'un handicap sont évidemment des sujets essentiels. À l'heure actuelle, on comptabilise près de 96 000 contrats aidés conclus, au titre de 2017, par les associations. Ce chiffre n'est pas stabilisé, les employeurs devant transmettre leurs dossiers en fin d'année. Une politique de l'emploi efficace doit s'appuyer sur le renforcement des politiques de formation et d'accompagnement ciblé, lesquelles permettent des taux de retour à l'emploi durable plus significatifs pour les bénéficiaires. Ma collègue ministre du travail, Muriel Pénicaud, a confié une mission à M. Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, visant à mobiliser les acteurs de l'insertion autour de nouvelles solutions, au service du parcours de chacun et en particulier de ceux qui sont aujourd'hui les plus largement exclus de l'accès au marché du travail. Les propositions vont lui être remises sous peu. C'est donc une politique efficace de lutte contre le chômage qui est engagée. En parallèle, le Premier ministre m'a demandé de préparer une nouvelle stratégie pour le quinquennat en faveur de la vie associative. Cette stratégie doit être en harmonie avec le plan pour l'économie sociale et solidaire. Après une réunion de lancement en décembre dernier, avec notamment les acteurs associatifs, les premières réunions de travail se tiennent aujourd'hui même.

Plus généralement, la mise en oeuvre d'une étude d'impact contradictoire sur l'évolution des financements publics aux associations, sur les actions qu'elles mènent et sur les conditions d'emploi de leurs salariés permettrait de renouer le lien entre l'État,

Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention, et celle du Gouvernement, sur les questions que se posent de nombreux maires au sujet du fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour les prochaines rentrées scolaires. Malgré les nombreuses hésitations et plusieurs changements de cap ces dernières années en matière d'organisation du temps scolaire, la semaine de quatre jours et demi reste la règle. Dans nos territoires, les élus sont confrontés à de nombreuses difficultés, principalement financières, pour maintenir la semaine de quatre jours et demi. Bien entendu, cette situation a des répercussions sur la pertinence, mais aussi sur la qualité des activités périscolaires qui sont proposées aux élèves. Ainsi, le régime dérogatoire avec l'organisation de la semaine scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est bien souvent sollicité auprès des directions académiques. Si l'organisation du temps scolaire répond à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école, les élus doivent pouvoir délibérer en amont pour faire des choix en adéquation avec leur budget communal. C'est pourquoi le fonds de soutien au développement des activités périscolaires est indispensable. Des communes continuent à mettre en oeuvre la réforme. À cette fin, elles ont organisé des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Les marges de manoeuvre budgétaires sont limitées, voire quasi inexistantes aujourd'hui. Il est donc indispensable d'avoir des certitudes et d'obtenir les informations nécessaires de la part du Gouvernement afin de préparer le budget communal. Dans notre département de la Loire, les communes ont jusqu'au 10 février 2018 pour se prononcer sur l'organisation du temps scolaire. En conséquence, les élus ont besoin de connaître les modalités pratiques et les montants des aides prévues dans le cadre de ce fonds de soutien spécifique.

Là où les communautés éducatives et les communes sont satisfaites de l'organisation qu'elles avaient, elles ont pu continuer à fonctionner selon les mêmes modalités. Le fonds a été perpétué pour elles. Là où a émergé un consensus local en faveur d'une autre organisation, une dérogation aux cadres existants a été possible.

À l'issue des différentes périodes de concertation qui se sont succédé, des consensus locaux ont émergé pour la prochaine rentrée. Nous voyons progressivement certaines communes passer à quatre jours et d'autres rester à quatre jours et demi. Les intentions du Gouvernement en matière d'organisation du temps scolaire sont donc très claires. Les modalités pratiques et financières de préparation de la prochaine rentrée sont stabilisées et transparentes. En effet, il est très important que les parties prenantes à l'échelon local disposent de cette visibilité pour préparer sereinement la rentrée. Les communes qui conserveront une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées par semaine, ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées, continueront à percevoir les aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires.

Sur le plan budgétaire, le Gouvernement tient ses engagements. Les acomptes ont été versés aux communes éligibles il y a quelques semaines et les crédits nécessaires ont été prévus en loi de finances pour 2018. Les montants, tels que définis par l'arrêté du 17 août 2015 fixant les taux des aides du fonds de soutien au développement des activités périscolaires, soit 50 euros pour pour le taux du montant forfaitaire et 40 euros pour le taux de la majoration forfaitaire, sont maintenus. Nous n'oublions pas le besoin de simplifier chaque fois que possible les procédures de gestion, comme l'ont demandé les communes. Une mesure d'allégement a été mise en place pour la gestion 2017-2018 à la suite de la modification du décret du 17 août 2015. Ainsi, les acomptes de la campagne 2017-2018 ont été versés, sans demande préalable,

Le drame vécu par les réfugiés ne peut naturellement nous laisser indifférents. Il nous appartient de nous mobiliser pour rechercher les meilleures conditions d'accueil. Tous les réfugiés irakiens ne présentent pas un faible niveau de qualification.

d'un des systèmes éducatifs les plus performants du Moyen-Orient. Le taux de scolarisation y était excellent, l'école y était gratuite et obligatoire et la scolarisation des filles y atteignait un bon niveau. L'enseignement secondaire y offrait aussi des formations de qualité, particulièrement dans les établissements d'enseignement scientifique et technologique. Le pays comptait plus d'une vingtaine d'universités publiques ainsi que des facultés privées. Malheureusement, une fois en France, les réfugiés irakiens rencontrent des difficultés à faire valoir leurs diplômes et leurs expériences acquises. Actuellement, il est important de noter qu'il n'existe pas de principe juridique d'équivalence entre les titres et les diplômes obtenus en Irak et les diplômes français. Seule une attestation de reconnaissance d'un certain niveau d'études atteint par comparaison au système français peut être obtenue. Par ailleurs, selon que le diplôme porte sur l'exercice d'une profession réglementée ou non réglementée, la procédure n'est pas la même. Par exemple, les détenteurs d'un diplôme de docteur en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie, ou d'un diplôme de sage-femme, obtenu en Irak, ne peuvent exercer sur le territoire français qu'après avoir eu l'autorisation de l'ordre ou du conseil national compétent, ce qui est d'ailleurs logique. Ces procédures de reconnaissance et de comparabilité sont parfois longues, compliquées et difficilement accessibles aux bénéficiaires d'une protection internationale.

de faire évoluer notre système et de faciliter la reconnaissance des titres et diplômes universitaires irakiens de qualité. Cet enjeu vaut d'ailleurs pour d'autres États que je n'ai pas cités. Le Gouvernement envisage-t-il d'instaurer une convention bilatérale avec ce pays, qui dispose aujourd'hui d'institutions

dispose qu'Israël est « l'État-nation du peuple juif » avec Jérusalem pour capitale et l'hébreu comme seule langue officielle. Il précise également que le droit à l'autodétermination est réservé au seul peuple juif. La langue arabe, parlée par au moins 20 % d'Israéliens issus de la minorité arabe, perdrait ainsi son statut et ne serait plus une des langues officielles de l'État. Enfin, une disposition de ce définit et légalise une ségrégation ethnique en autorisant un groupe d'une même religion à vivre en communauté, séparé des autres. Cette mesure permet l'établissement de communautés exclusivement juives. ce projet de loi risque d'aggraver grandement le statut de la minorité arabe des citoyens d'Israël, mais il va à l'encontre des principes démocratiques et institutionnalise des discriminations raciales.

En effet, la résolution de cette situation passe par la mise en place des deux États. Toute mesure susceptible de créer des discriminations entre citoyens juifs et arabes en Israël constituerait un obstacle supplémentaire sur cette voie. Vous connaissez, en outre, la position constante de la France au sujet de Jérusalem.

l'amie du peuple palestinien, comme elle est l'amie du peuple israélien, et ce lien d'amitié nous permet aussi de dire les choses très franchement. Ainsi, en accueillant

remettre en cause les relations internationales et les règles internationales que les pays se donnent. La

Après avoir connu l'emprisonnement pendant sept longues années, il fait face, une nouvelle fois, à une décision arbitraire. Salah Hamouri a été arrêté chez lui au petit matin le 23 août dernier et placé en détention administrative pour six mois sur ordre du ministère de la défense israélien. Or la détention administrative ne permet ni à Salah Hamouri ni à ses avocats d'avoir accès à son dossier, pas plus que de connaître les raisons ou les preuves supposées qui ont conduit à son incarcération. Vous le savez, la détention administrative est contraire au droit international. Elle a été utilisée de manière systématique par plusieurs régimes répressifs pour contourner la voie judiciaire et priver des opposants politiques, des résistants pacifiques et, plus largement, de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens de la protection légale à laquelle ils ont droit. Emprisonné sans pouvoir se défendre ni savoir ce qu'on lui reproche : telle est la situation de notre compatriote depuis 147 jours ! Depuis cet été, la France n'est pas restée inactive. Le Quai d'Orsay a dénoncé « l'utilisation abusive et systématique de la détention administrative La France a « espéré » sa libération avant de la « demander » en décembre dernier. Nous savons aussi que le Président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué la question lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Paris, le 10 décembre dernier, comme il l'a écrit à de nombreuses associations. Pourtant, depuis lors, la situation de notre compatriote ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Le 31 décembre dernier, par mesure de rétorsion, l'administration pénitentiaire a déplacé notre compatriote de la prison du Neguev à celle de Megiddo, à la suite de l'interview qu'il a accordée national. Cette situation est inacceptable, et la France ne peut l'accepter. Chaque jour supplémentaire que Salah Hamouri passe en prison est un jour de moins passé avec sa femme, son fils et sa famille, qui ont déjà trop souffert. Chaque jour supplémentaire est une offense faite à la France et aux droits de l'homme les plus élémentaires. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est simple et directe : quels gestes nouveaux notre diplomatie va-t-elle accomplir pour obtenir enfin la libération immédiate de notre jeune compatriote ?

six mois. Nous suivons cette situation avec la plus grande attention. Ce n'est pas une clause de style : j'ai eu à en connaître personnellement à plusieurs reprises. Naturellement, Salah Hamouri bénéficie, comme l'ensemble des Français emprisonnés à travers le monde, de la protection consulaire, conformément à la convention de Vienne. Il a pu recevoir à ce titre plusieurs visites de nos autorités consulaires depuis le début de sa détention. La dernière en date, effectuée par notre consul à Haïfa, jours. Il est vrai que le régime de détention administrative est d'une nature particulière. Il ne permet pas à Salah Hamouri d'avoir accès aux charges retenues contre lui ; nous ne les connaissons pas non plus. J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir à l'ambassadrice d'Israël en France pour lui redire tout notre attachement à la résolution de cette situation. La position de la France à ce sujet est claire, et je la rappelle : nous condamnons l'utilisation abusive de la détention administrative, qui porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense. Tel est le message que nous ne cessons de passer. Dans ces conditions, nous continuons à demander le plein respect des droits de notre compatriote et à espérer sa libération rapide. Dans l'immédiat, et de manière urgente, nous réitérons notre souhait que sa famille

la formation professionnelle continue des pâtres. Mais, en la matière, l'enjeu est également la transition écologique et solidaire, madame la secrétaire d'État, puisque les bergers saisonniers sont des acteurs majeurs du pastoralisme, activité vitale pour la sauvegarde de la biodiversité dans nos montagnes.

souhaitent accéder à la formation professionnelle continue, mais ils en sont exclus, alors même que leurs employeurs cotisent à un organisme paritaire collecteur agréé : le Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles, le FAFSEA. Cette exclusion par le fait que les droits associés aux contrats de travail pour ces travailleurs saisonniers, parmi lesquels celui de l'accès à la formation, ne sont reconduits que lorsque ces contrats sont renouvelés, à chaque nouveau début de saison. De fait, durant les périodes d'intersaison, alors que les travailleurs seraient généralement disponibles, ils ne peuvent activer ces droits associés, car ils ne sont précisément plus sous contrat. Pour pallier cette difficulté, le FAFSEA a bien proposé aux employeurs de salarier leurs pâtres quelques jours avant la montée en estive afin de leur permettre de se former avant leur prise de poste.

qui, en raison des particularités de leur métier, ne peuvent être disponibles pour suivre une formation pendant la durée de leur contrat de travail saisonnier. Vous nous faites part du fait que, durant les périodes d'intersaison, les pâtres n'étant plus sous contrat de travail, ils ne peuvent bénéficier d'aucun programme de formation, alors même que leurs employeurs

lequel prévoit un dispositif de formation particulier destiné aux salariés occupant un emploi saisonnier et ne pouvant se libérer pour une action de formation au cours de leur contrat. Cet article permet, sous certaines conditions, à l'employeur d'un salarié saisonnier qui s'est engagé à reconduire son contrat pour la saison suivante, de conclure un contrat de travail à durée déterminée pendant la période d'intersaison. Ce contrat a pour objet de permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise, et sa durée est égale à celle qui est prévue pour l'action de formation. l'organisme paritaire collecteur agréé, ou OPCA, compétent. Nous prenons toutefois acte du fait que cette solution pratique proposée à l'heure actuelle par le FAFSEA ne permet pas de répondre aux enjeux de la formation professionnelle des pâtres : je vous remercie d'avoir attiré l'attention de Mme la ministre du travail sur ce point. Ses services se rapprocheront de ceux du FAFSEA pour étudier les pistes d'amélioration susceptibles d'être suivies. Par ailleurs, il convient de vous préciser que, lors des périodes d'intersaison, le pâtre, qui revêt le statut de demandeur d'emploi, a aussi la possibilité d'accéder à l'ensemble des dispositifs de formation dédiés aux salariés privés d'emploi, financés notamment par Pôle emploi et par les régions.

Malheureusement, certaines décisions récentes ont conduit à affaiblir les réseaux associatifs locaux. La plupart des associations subissent à la fois la baisse importante de leurs financements et la réduction du nombre des emplois aidés.

et des salariés souvent engagés. Leur importance est considérable sur un territoire comme le nôtre. Elles jouent un rôle de lien social fort, même lorsqu'elles sont directement concurrencées par le secteur marchand lucratif. La réduction des contrats aidés met en péril, par exemple, l'activité de l'association « Projets, échanges et développement » de Plougasnou, petite commune littorale du Finistère, en raison de la non-reconduction à son poste de la secrétaire comptable. L'activité de l'association de développement des circuits courts alimentaires par la distribution de paniers bio et la mise en relation des producteurs et des consommateurs de Brest est compromise par la mise en danger de trois des quatre salariés de cette structure. Je partage avec vous l'idée selon laquelle l'économie sociale et solidaire doit pouvoir changer d'échelle et passer un cap de développement. Les derniers signaux envoyés aux acteurs ne me semblent pourtant pas de nature à rassurer le monde associatif et le monde de l'économie sociale et solidaire. Avec le Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire, vous avez lancé quelques pistes en matière de développement. À ce jour, le monde associatif n'en demeure pas moins en attente d'un accompagnement fort de la puissance publique, non seulement en termes de moyens économiques, mais également en matière de sécurisation financière, ainsi, me semble-t-il, que de stabilisation de la politique économique en faveur des associations dont l'activité pourrait être compromise par la mise en concurrence de la commande publique ou par l'insécurité liée aux variations de subventions. Madame la secrétaire quelles sont vos intentions en matière de sécurisation de l'activité associative de notre pays ?

la diminution du nombre d'emplois aidés et la suppression de la réserve parlementaire auront des conséquences pour les associations. Toutefois, l'État agit sur plusieurs fronts pour les aider à fortifier leur assise économique et pour les rendre moins sujettes aux variations conjoncturelles, comme tel a pu être le cas ces dernières années avec les emplois aidés. Tout d'abord, le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, ou CITS, sera maintenu en 2018. Il représente un gain annuel de 500 millions d'euros pour les associations, qui en sont les principales bénéficiaires. des entreprises, le CITS sera relevé de deux points et converti en réduction pérenne de cotisations patronales afin d'encourager l'emploi et de consolider structurellement le modèle économique de toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Si l'on ajoute à cela l'effet du dispositif « zéro charge patronale pour le SMIC », lequel entrera en vigueur le 1 janvier 2019, c'est 1,4 milliard d'euros de marges de manoeuvre annuelles qui seront libérés au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

L'augmentation de cette ligne budgétaire est une demande récurrente des représentants associatifs depuis de nombreuses années. Nous travaillons actuellement à faire évoluer ce fonds vers un renforcement des dispositifs d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des associations de terrain, mais aussi de formation, voire d'expérimentation de dispositifs innovants ou d'installation de dispositifs éprouvés. Ce travail se fera bien entendu en concertation avec les réseaux associatifs, qu'ils soient nationaux, régionaux ou de proximité. Sur ce point, nous travaillons actuellement avec les opérateurs du dispositif local d'accompagnement, le DLA, afin qu'ils développent dans les plus brefs délais une offre de services spécifique en direction des associations ayant disposé ou disposant d'emplois aidés au titre de la période 2017-2018. De manière plus globale, le plan de développement de l'économie sociale et solidaire, que le Gouvernement souhaite impulser à partir de cette année, aura un impact direct sur les associations, lesquelles représentent plus de 80 % des entreprises du secteur. Enfin, puisque la

L'objet de cette concertation est précisément d'écouter spécifiquement les problématiques associatives pour les prendre en compte dans un plan de développement associatif, qui sera distinct, mais complémentaire, du plan de développement de l'économie sociale et solidaire.

je souhaite vous alerter sur les difficultés engendrées par la classification des cours d'eau et, plus généralement, sur les dérives liées à l'inflation des normes. La loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016 a fixé trois critères cumulatifs pour définir de manière claire un cours d'eau : ce doit être un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Or les directions départementales des territoires et l'Agence française pour la biodiversité surinterprètent ces critères en se référant à des éléments complémentaires élaborés par l'administration de votre ministère. Des écoulements se retrouvent alors injustement qualifiés en cours d'eau et, encore plus grave, en cas de doute, cette qualification est même devenue automatique ! Les règles applicables à un cours d'eau étant bien plus contraignantes et coûteuses, les conséquences sont graves pour les collectivités territoriales, et les contentieux les plus ubuesques se multiplient. À titre d'exemple, dans mon département du Territoire de Belfort, le maire de la commune de Lebetain a été condamné récemment à une amende de 500 euros avec sursis pour avoir procédé au nettoyage du lavoir communal. Que lui reproche-t-on ? Eh bien, d'avoir réalisé des travaux d'entretien imposés par la loi sans détenir le récépissé de déclaration de la DDT ! Seulement, pour obtenir ce récépissé, ce maire aurait dû débourser 27 000 euros pour constituer le dossier environnemental obligatoire. Dans le contexte actuel de baisse des concours financiers de l'État, cette commune de 450 habitants, dont le budget annuel de fonctionnement est de 235 000 euros, n'est évidemment pas en mesure de s'acquitter d'une telle somme. Notez d'ailleurs que ce montant lui est réclamé pour chaque entretien de l'édifice Cette opération de curage est pourtant indispensable pour prévenir les inondations. Ce maire a donc été condamné alors qu'il agissait dans le respect de son obligation générale de prévention des accidents naturels. C'est pourquoi je vous demande, madame la secrétaire d'État, de quelle manière vous entendez éclaircir juridiquement la classification des cours d'eau, qui pose beaucoup de problèmes dans le milieu rural. Quelles mesures sont-elles prises par le Gouvernement pour réduire les coûts obligatoires à la charge des collectivités en matière environnementale ? Enfin, comment orienter un maire de bonne foi,

Vous avez appelé mon attention sur la réglementation relative à l'entretien des cours d'eau et son articulation avec les responsabilités des élus. Votre question me permet, tout d'abord, de rappeler que les cours d'eau sont des écosystèmes fragiles qu'il faut impérativement préserver au travers d'un entretien adapté, permettant l'écoulement naturel des eaux. Cela est primordial pour éviter l'aggravation des inondations, à l'amont comme à l'aval. Afin de lever les incompréhensions qui subsistent sur le terrain, l'instruction du Gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l'identification des cours d'eau et à leur entretien a permis la diffusion de guides déclinés localement, à l'attention des propriétaires riverains de cours d'eau, sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour préserver les milieux aquatiques. Cet entretien, qui est une obligation, consiste en l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements et l'élagage ou recépage de la végétation des rives. Il n'est soumis à aucune procédure préalable. Les fossés sont, quant à eux, des ouvrages artificiels dont le maintien en bon état de fonctionnement n'est pas non plus soumis à une procédure préalable. Les interventions sur les cours d'eau, qui vont au-delà de cet entretien, peuvent avoir des impacts importants sur les écosystèmes et sur les autres riverains. Elles sont donc soumises à une procédure préalable pour en vérifier le bien-fondé et les potentiels inconvénients. Les agents de la police de l'environnement, dont ceux de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, sont chargés de veiller à la bonne application de la réglementation. Leurs actes sont soumis au contrôle du juge. Dans l'exemple que vous citez, la réalisation de travaux sans titre a abouti à une condamnation pénale du maire par le tribunal de police Selon les informations portées à ma connaissance, les services de l'AFB ont alerté à plusieurs reprises l'élu sur les conséquences de l'opération et sur la nécessité de déposer une déclaration au titre de la loi sur l'eau, à un coût bien moindre que celui indiqué. Enfin, depuis le 1 janvier 2018, la compétence dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la GEMAPI, est une compétence obligatoire des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, à fiscalité propre.

Les dispositions du code de l'environnement et celles du code général des collectivités territoriales ne présentent donc pas de contradictions. Sachez que le Gouvernement oeuvre pour que les collectivités locales disposent des outils adaptés pour prendre en compte les enjeux de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à la bonne échelle et selon l'organisation la plus adaptée.

conscience de la nécessité de le préserver. Reste que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, ou alors nous ne vivons pas tout à fait dans la même France. Le milieu rural souffre de ces difficultés

La pollution de l'air est en effet devenue la troisième cause de mortalité dans notre pays. Cette situation ne peut évidemment que nous préoccuper. Ces annonces ont eu lieu le lendemain même du jour où le Président de la République confirmait les engagements de l'État vis-à-vis du Lyon-Turin lors du sommet franco-italien de Lyon. Le Lyon-Turin se trouve ainsi au coeur des enjeux énergétiques et environnementaux grâce à l'ambition du report du transport de marchandises de la route vers le rail. L'ambition du département de Savoie a toujours été d'enlever le trafic ferroviaire de marchandises qui longe le lac du Bourget, premier lac naturel de France, et traverse les agglomérations d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Or, dans le même temps, le volume de marchandises transportées par la route de la France vers l'Italie a progressé de 1 % par an entre 2006 et 2016. Alors qu'entre la France et l'Italie le volume de marchandises transportées par le rail n'arrive pas à progresser faute d'infrastructures et de services adaptés, dans le même temps le volume de marchandises transportées par le rail entre la Suisse et l'Italie a progressé de 5 % par an. Ainsi, en 2016, le trafic de marchandises entre la France et l'Italie a été de 40 millions de tonnes, soit identique à celui entre la Suisse et l'Italie. En revanche, malgré la hausse du trafic, la Suisse est passée pour la première année en dessous de un million de poids lourds, alors que, avec presque trois millions de poids lourds, le trafic routier continue de progresser en France. Or l'AFA, l'autoroute ferroviaire alpine, qui devait traduire l'ambition du report modal de la France, soit le transfert de un million de poids lourds, ne permet d'atteindre aujourd'hui qu'un peu moins de 3 % de cet objectif, qui ne bénéficie d'aucune véritable impulsion politique. L'appel d'offres en cours concernant la plateforme dite de « l'est lyonnais » a été décidé en 2009 et n'est toujours pas attribué. Ainsi, la société MSSA, située dans la vallée de la Tarentaise, qui a un besoin impératif pour ses matières dangereuses de 500 unités de transport par an, ne peut bénéficier de la part de l'AFA que d'une capacité de 400 unités. À l'heure où le Gouvernement souhaite afficher des ambitions fortes et s'engager dans une dynamique volontariste, encore convient-il que des mesures concrètes et urgentes soient prises à l'instar des politiques du transport de marchandises chez nos voisins européens. pourriez-vous indiquer quels engagements le Gouvernement compte prendre pour être à la hauteur de ce défi, qui est autant un défi économique qu'écologique ?

Ils ont pu constater combien les problématiques de transport routier, de report modal et de qualité de l'air sont essentielles dans l'arc alpin. La mise en service du tunnel ferroviaire Lyon-Turin a pour objectif de limiter la congestion et les nuisances sonores et atmosphériques liées au trafic routier de poids lourds, d'améliorer le cadre de vie des riverains, en particulier dans la vallée de la Maurienne, et de lutter contre le changement climatique. À titre d'exemple, l'ouverture du tunnel permettra d'économiser en moyenne trois millions de tonnes de CO2. Le sommet franco-italien du 27 septembre dernier a d'ailleurs confirmé l'engagement des deux États en faveur de la réalisation de cette nouvelle infrastructure, qui est centrale pour la stratégie de report modal dans la traversée des Alpes. Le report modal repose également sur une politique volontaire pour valoriser l'autoroute ferroviaire alpine, qui permet dès maintenant d'offrir une alternative au transport routier de marchandises. Le trafic de l'autoroute ferroviaire alpine est en progression de plus de 25 % pour l'année 2017 et pourrait dépasser ainsi les 35 000 poids lourds transportés. Après la France en 2010, l'Italie a ratifié, le 22 novembre 2017, l'accord du Luxembourg, signé en 2009, permettant la mise en concession de ce service. Le 1août dernier, un avis de concession a été publié au de l'Union européenne. La procédure binationale devrait donc aboutir à une mise en concession courant 2019. Dans ce contexte, le protocole conclu en 2014 avec la collectivité d'Aiton permet effectivement de garantir la mise à disposition du terminal français nécessaire à la continuité du service de ferroutage indispensable au développement de la société que vous avez citée.

que l'enthousiasme et l'engagement de M. le ministre Hulot, dont je ne conteste absolument pas la volonté, puissent se traduire dans les faits. La société que j'ai citée comme exemple sera une bonne illustration de la capacité que l'on a

Comme vous le savez, ce train a été classé en 2015 parmi les trains d'équilibre du territoire, puisqu'il n'existe pas d'offre ferroviaire alternative entre l'Île-de-France et le département des Hautes-Alpes. Or force est de constater que les difficultés de réservation pour le Paris-Briançon sont récurrentes, alors que ce mode de transport correspond à un réel besoin et répond aux attentes, notamment des touristes franciliens. Pour les dernières vacances de fin d'année, la réservation a été ouverte deux semaines avant les premiers départs. À ce jour, il est impossible de réserver un billet pour les vacances de printemps, qui débuteront le 14 avril, puisque ce train n'apparaît même pas sur le site de la SNCF. Si l'on voulait dissuader les voyageurs d'utiliser le Paris-Briançon, on ne s'y prendrait pas autrement Je tiens à préciser que, en période de vacances, ce produit est majoritairement utilisé par les familles, qui peuvent ainsi accéder aux stations de sports d'hiver de Serre-Chevalier ou de Vars-Risoul, par exemple, sans rupture de charge avant la gare d'arrivée, ce qui n'est pas négligeable, notamment pour les personnes voyageant avec de jeunes enfants. Madame la secrétaire d'État, face aux difficultés récurrentes de réservation et en l'absence de dispositions efficaces de la part de SNCF Mobilités, je vous serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer quelles dispositions ont été prises pour que la SNCF honore son contrat avec l'État. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire.

L'ouverture tardive des ventes a résulté d'une difficulté technique à tracer des sillons exploitables pour les trains de nuit et compatibles avec les différentes plages de travaux opérés par SNCF Réseau. Afin de régulariser au plus vite les difficultés rencontrées pour les périodes des fêtes de fin d'année 2017 et la haute saison hivernale 2018, la ministre chargée des transports a demandé à SNCF Réseau et SNCF Intercités de trouver des solutions permettant de garantir la circulation d'un maximum de trains durant ces périodes primordiales pour les Hautes-Alpes. Ce travail a porté ses fruits, puisque, à de très rares exceptions, tous les trains ont été ouverts jusqu'au 16 mars. Par ailleurs, malgré l'ouverture tardive de la vente des billets, cette offre de transport a été plébiscitée par les vacanciers, et les trains ont affiché complet pour les vacances de Noël. C'est également le cas pour les week-ends de départ des vacances d'hiver des académies franciliennes, les vendredi 16 et samedi 17 février, et le vendredi 23 février. Cela prouve l'importance de ce service pour l'économie touristique des Hautes-Alpes et du Briançonnais en particulier. Enfin, afin de pallier l'arrêt de la pointe neige, dispositif qui était extrêmement coûteux ramené au voyageur, la ministre chargée des transports a demandé que la composition des trains soit renforcée pour les week-ends des vacances de février pour offrir des places supplémentaires nécessaires à la bonne desserte de ce territoire. La parole

par une voie ferrée unique et par une autoroute qui n'a jamais été terminée. Je regrette que la destination Hautes-Alpes ne bénéficie pas d'une desserte ferroviaire qui, à défaut d'être performante, soit au moins opérationnelle comme c'est le cas pour d'autres territoires de montagne.

Plusieurs villes de province, notamment Aurillac, Brive, Castres, Agen, sont desservies au niveau aérien par ces lignes dans le cadre d'obligations de service public, les OSP, bénéficiant du concours financier de l'État, qui s'ajoute aux subventions apportées par les collectivités locales. Ces concours financiers publics représentent jusqu'à deux tiers du coût du fonctionnement de ces lignes, le prix payé par les passagers n'étant pas, pour autant, très abordable. Malgré ces efforts financiers considérables, il s'avère que le fonctionnement quotidien de ces lignes, considérées comme concédées à la compagnie Hop !, filiale d'Air France, est de plus en plus problématique- c'est un euphémisme En effet, le service se dégrade considérablement, avec des retards extrêmement fréquents et des annulations de vols, pour des raisons dites techniques. La situation a clairement empiré depuis le mois de septembre, avec souvent plusieurs annulations de vols chaque semaine. Cela est d'autant plus problématique que, sur ces lignes, il n'y a déjà aucun vol les samedis, dimanches matin et jours fériés. Une telle dégradation du service public est inacceptable et ne fait qu'aggraver la fracture dont pâtissent des territoires déjà très très excentrés, mettant en danger leur vie économique. Madame la secrétaire d'État, quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier à cette situation devenue intolérable et contraindre la compagnie Hop !, filiale d'Air France, à assurer enfin un service public digne de ce nom ? La parole

réponds au nom de la ministre chargée des transports, qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. La desserte aérienne des territoires, notamment des plus enclavés, est un enjeu majeur de la politique française des transports. La ministre chargée des transports suit d'ailleurs avec beaucoup d'attention la situation actuelle des liaisons opérées par la compagnie Hop Cette dernière, issue de la fusion de trois compagnies régionales du groupe Air France, a récemment été confrontée à un déficit du nombre de pilotes, lié à une évolution des carrières de ces derniers au sein du groupe, et à une succession de pannes techniques sur ses appareils de type ATR 42. De septembre à décembre 2017, certaines lignes ont ainsi connu un nombre d'annulations exceptionnel, allant jusqu'à diminuer de 10 % le nombre de vols réalisés par rapport à la même période en 2016. Sur l'ensemble de l'année 2017, près de 6 % des vols reliant Paris à Aurillac, Brive, Castres et Agen ont été annulés pour des causes directement imputables à la compagnie, alors que la tolérance en termes d'obligations de service public ne s'élève qu'à 3 %. La qualité de service et la ponctualité des vols réalisés par la compagnie se sont en outre trouvées affectées par d'autres facteurs, tels que les travaux engagés à l'aéroport de Paris-Orly, nécessaires à la mise en conformité de la plateforme aux règles européennes de sécurité aérienne. Les retards et les annulations que connaissent les vols du réseau opéré par Hop ! ne sont pour autant acceptables ni pour les passagers ni pour les territoires concernés. Il n'est pas admissible qu'ils puissent remettre en cause l'amélioration de l'équilibre économique et l'augmentation de trafic globalement observées en 2017 sur ces liaisons d'aménagement du territoire. La Direction générale de l'aviation civile est mobilisée pour accompagner les territoires à faire valoir auprès de la compagnie le préjudice économique subi, en la pénalisant financièrement dans les conditions prévues par les conventions signées. Mais il est avant tout primordial que Hop ! retrouve au plus vite des conditions opérationnelles plus robustes. La compagnie a assuré la ministre chargée des transports de sa volonté de rester un acteur majeur du désenclavement et de l'aménagement des territoires et lui a confirmé avoir mis en place un plan d'actions spécifique de maintenance préventive afin de limiter les indisponibilités techniques de ses appareils. Hop ! accélère également les recrutements et les formations de pilotes pour faire face aux nombreux départs et respecter ses engagements dans le cadre des délégations de service public en vigueur. Le ministère chargé des transports continuera de porter une attention particulière à ce sujet et demandera un compte rendu régulier à Hop ! des actions menées et de leur impact concret sur le fonctionnement quotidien des lignes concernées,

a pour ambition d'encourager la revitalisation des centres-bourgs des villes moyennes. Ces mesures vont dans le bon sens tant il y a à faire dans ce domaine ; elles semblent cependant donner la priorité aux villes moyennes et exclure les communes les plus rurales de notre territoire. En effet, seules les communes ayant un « rayonnement régional » ou toutes celles jouant un rôle de « centralité pour leur bassin de vie » seront éligibles au financement. Ainsi, dans les faits, les villes de moins de 8 000 habitants auront peu de chances d'y avoir accès. C'est fort regrettable, par exemple pour mon département, la Mayenne, où 44 % des 255 communes comptent moins de 500 habitants et où seules cinq communes ont plus de 8 000 habitants. Peut-être considérez-vous que cette strate a déjà bénéficié de l'appel à manifestation d'intérêt « centres-bourgs » en 2014 ? Je vous informe que, à l'époque, aucun dossier présenté par mon département n'avait été retenu. La situation devient donc préoccupante pour ces communes rurales : désengagement de l'État, baisse des dotations et des ressources financières, dépossession progressive des compétences- eau et assainissement, urbanisme, carte d'identité -, fermeture des commerces de proximité, tels que les cafés, les supérettes, les salons de coiffure, les bureaux de poste

Les élus locaux et les habitants sont attachés à l'entité communale traditionnelle, parce que celle-ci crée du lien social et favorise la proximité. Les élus se battent pour préserver leur territoire

le Gouvernement confirme et conforte le soutien aux projets d'investissement dans les communes et les intercommunalités rurales. Il promeut également toute forme de coopération locale entre différents territoires, en vue d'instaurer une plus grande cohésion au sein des bassins économiques et de vie.

Ces contrats de ruralité ont pour objet d'encourager les projets des communes rurales au sein des EPCI et des PETR. Cette première génération de contrats sera mise en oeuvre jusqu'en 2020, avec un engagement de cofinancement de la DETR et de la DSIL dans le budget quinquennal de l'État. En 2018, afin de soutenir les capacités d'investissement, la DETR est maintenue à hauteur de plus de 1 milliard d'euros, soit le montant financier le plus élevé de l'histoire de cette dotation, en augmentation de 50 millions d'euros par rapport à 2017. La DSIL se chiffre, quant à elle, à 615 millions d'euros, ce qui permet d'assurer notamment le cofinancement de projets prêts à démarrer en 2018 et inscrits dans les plans d'action des contrats de ruralité. De plus, avec l'engagement, cette année, du plan Action coeur de ville, annoncé les 14 et 15 décembre dernier, des communes centres d'un bassin de vie à dominante rurale exerçant une fonction de « ville moyenne » seront accompagnées et soutenues financièrement dans leur projet de requalification de leur centre-ville, au bénéfice de l'attractivité et des habitants du territoire. Par ailleurs, si, dans un objectif de maîtrise des finances publiques, l'État contractualisera avec les 340 plus grandes collectivités afin que la hausse de leurs dépenses de fonctionnement n'excède pas les 1,2 % par an, il en découle que 99 % des collectivités ne seront pas concernées par cette contractualisation, parmi lesquelles figurent toutes les communes rurales. Poursuivre les efforts majeurs engagés ces dernières années en faveur des ruralités dans tous les domaines reste également une priorité. En particulier, la couverture numérique des territoires par les réseaux fixes et mobiles est une priorité du Gouvernement. Vous connaissez les annonces récentes Je rappelle les ambitions du Président de la République, qui, en juillet dernier, a annoncé son souhait d'accélérer les programmes en cours, en fixant pour objectif l'accès à du bon haut débit pour tous les Français dès 2020. Le Gouvernement souhaite aussi travailler, en coconstruction avec les élus, à trouver de

qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues » par le décret, d'autres membres de la famille ou une pacsée. Il semble que la plupart des caisses d'assurance maladie méconnaissent les effets de ce décret et indiquent aux conjoints des assurés sociaux, à leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par un PACS que, à défaut d'être eux-mêmes assurés, ils sont soumis au critère de résidence et, donc, au délai de carence de trois mois pour pouvoir être affiliés à la sécurité sociale.

vous avez appelé l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur des difficultés d'application du décret du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie, dite Vous signalez des situations dans lesquelles des personnes arrivées en France pour rejoindre leur conjoint, déjà assuré social, se voient opposer un délai de carence de trois mois pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé. La protection universelle maladie, entrée en vigueur depuis le 1 janvier 2016, garantit à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Pour l'ouverture du droit à la prise en charge de ces frais, le critère de stabilité est réputé satisfait lorsque la personne présente un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Pour autant, et comme vous l'indiquez, je vous confirme que ce délai de trois mois ne s'applique pas aux conjoints, concubins et partenaires de pacte civil de solidarité qui rejoignent ou accompagnent, pour s'installer en France, un assuré y séjournant lui-même de façon stable et régulière. Ces personnes bénéficient donc de la prise en charge de leurs frais de santé sans délai de carence, à la condition qu'elles soient en situation régulière au regard de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et du droit d'asile. suite de votre alerte, les services du ministère des solidarités et de la santé se sont rapprochés de ceux de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour lui demander que cette dernière effectue un rappel à la règle dans les plus brefs délais aux caisses de son réseau pour garantir la bonne application de cette disposition. La parole

En effet, l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté évoque, à l'occasion de l'élaboration de son projet régional de santé, la fermeture du centre 15 du SAMU 58 pour le transférer au centre hospitalier universitaire de Dijon. Cette annonce inquiète énormément la population, qui craint que cette décision n'ait un impact direct sur la prise en charge des patients nivernais. Je tiens à rappeler que la Nièvre est un département rural, touché par une désertification médicale galopante, alors même que sa population est particulièrement fragile en raison de son vieillissement. Comme vous le savez, le centre 15 gère plusieurs missions : les urgences vitales, mais aussi les missions de conseil aux patients. Les conseils représentent d'ailleurs une part importante de l'activité, surtout pour les personnes isolées. isolées. Du fait d'un plus grand nombre d'appels sur la plateforme régionale, qui, je vous le rappelle, devrait gérer huit départements, il y a de grands risques d'abandons d'appels sans pouvoir identifier les appelants ou encore un repli systématique des patients vers les structures d'urgence des hôpitaux déjà surchargées. Cette décision aurait également un impact sur les liens de proximité tissés au fil des années avec certains personnels médicaux, notamment dans le Morvan et le Nivernais central. Au-delà de la situation propre aux médecins, ce transfert poserait la question du devenir des assistants de régulation, qui sont les premiers interlocuteurs des appelants. Plus généralement, la question de la présence médicale dans nos départements ruraux devient de plus en plus cruciale. très nombreuses communes, dans la France entière, sont confrontées à un déficit dramatique de médecins et de spécialistes, tant libéraux qu'hospitaliers. Dans les cinq ans à venir, la Nièvre sera le département le plus touché par le départ à la retraite de généralistes. S'agissant des spécialistes, le département souffre également d'un manque criant de personnels dans certaines spécialités telles que la néonatologie, la pédopsychiatrie ou encore la psychomotricité. Or le droit d'être soigné constitue le premier des services que la collectivité doit rendre à ses concitoyens. L'égalité des soins constitue l'une des déclinaisons du principe d'égalité, qui est l'un des piliers de notre devise républicaine. Dans ce contexte, il est inimaginable d'envisager la disparition d'un service médical dans ce département. Une telle décision apparaîtrait comme un désengagement supplémentaire de l'État. Aussi quelles mesures

Cette question est, vous le savez, l'une des priorités de Mme Buzyn, qui a annoncé, le 13 octobre dernier, aux côtés du Premier ministre, un plan pour renforcer l'accès territorial aux soins. Dans le cadre des plans régionaux de santé, nous souhaitons améliorer l'accès aux soins de différentes façons. Votre question porte plus particulièrement sur le département de la Nièvre, notamment sur le transfert du centre 15 de la Nièvre, qui est en effet prévu dans le futur plan régional de santé.

dans la Nièvre. La région a une solide expérience. Cette organisation est d'ores et déjà en place en Franche-Comté où le centre 15 du CHU de Dijon assure avec efficacité la régulation des appels du 15 des quatre départements franc-comtois : le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. Cette régulation téléphonique au travers d'une plateforme travers d'une plateforme unique nous permet de redéployer sur le terrain les urgentistes, ressource particulièrement rare dans la Nièvre, dans les services des urgences du territoire, donc auprès des malades.

Se pose uniquement la question de l'organisation en nuit profonde, de vingt-deux heures à neuf heures du matin, des services d'urgence, avec une fermeture éventuelle sur un créneau à déterminer selon la réalité de l'activité de chaque site. Le ministère des solidarités et de la santé soutient la demande du préfet concernant le besoin d'un hélicoptère civil. Vos inquiétudes sont parfaitement légitimes. Actuellement, l'ARS travaille à améliorer globalement la desserte en transports sanitaires héliportés de toute la région. Nous souhaitons intensifier le recours aux moyens héliportés actuellement disponibles sur le territoire régional, et ce afin de libérer du temps pour les équipes médicales au sol. Cela passera par la définition d'une doctrine régionale d'emploi des moyens héliportés et une gestion mutualisée des appareils disponibles pour que ce soit bien, à chaque instant, l'appareil le mieux placé qui intervienne indépendamment de son site de rattachement. Monsieur le sénateur, j'espère avoir pu lever certaines de vos inquiétudes ; Mme la ministre des solidarités et de la santé pourra vous rassurer sur l'ensemble des points évoqués lors de sa visite dans votre département au début du mois de février pour les états généraux de la santé. La parole

Cette solution techniquement possible permettrait de renforcer l'attractivité du centre hospitalier de Nevers et constituerait de ce fait un élément de réponse à la difficulté de recruter des médecins. Aujourd'hui, il manque plus de cinquante médecins dans les effectifs de l'hôpital. Par ailleurs, permettez-moi d'insister encore sur les grandes difficultés dans lesquelles se trouvent les Nivernais pour accéder certains services indispensables. Prenons l'exemple des femmes enceintes. Au mois de décembre dernier, la population a vu la fermeture précipitée de la maternité de Cosne-sur-Loire après celle des maternités de Decize et de Clamecy. Aujourd'hui, sur un département de plus de 7 000 kilomètres carrés, nous n'avons qu'une maternité. Nous Nous sommes loin des objectifs de garantir à la population un accès, en moins de trente minutes, à une structure d'urgence. Le projet de suppression des urgences de nuit au centre

très fortement sollicités. Les pompiers constituent souvent le dernier recours sur nos territoires. Il paraît donc essentiel, au regard de notre démographie médicale déficitaire, de mettre rapidement en place une étude identifiant les risques de n'avoir personne sur certaines zones géographiques. Enfin, il faut tenir compte de la spécificité des territoires ruraux auxquels appartient le département de la Nièvre pour définir d'autres critères que ceux qui sont habituellement exigés par l'agence régionale de santé en vue de maintenir des activités de soins.

Mme la ministre des armées. « Jeunesse. L'âge du possible », écrivait Ambrose Bierce. Si cette étape de la vie est marquée du sceau de l'insouciance, elle n'en demeure pas moins importante, tant par les expériences, les découvertes que par les décisions qui en résultent. Toutefois, la situation de certains jeunes de notre pays demeure aujourd'hui préoccupante : chômage encore trop élevé, précarisation liée à un faible pouvoir d'achat, perte de repères. Il devient urgent de mettre en oeuvre une politique publique résolument ambitieuse pour cette génération. Aussi, parallèlement aux réformes économiques et sociales envisagées, le service national universel constituerait un tremplin d'émancipation et de solidarité, ce creuset de la cohésion nationale. En outre, les armées permettraient de recréer ce lien de confiance entre la République et la Nation. Elles ont ainsi un rôle majeur. Or, madame la secrétaire d'État, le parcours citoyen, tel qu'il a été dernièrement présenté par les députés, ne demeure pas satisfaisant sur la forme, et le fond et ne serait pas à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, la question de la durée est au coeur des débats. Un mois, initialement envisagé par le Président de la République, puis, désormais, une semaine par an paraissent insuffisants. En effet, cette durée ne permettrait pas de sensibiliser correctement les intéressés aux règles civiques et républicaines, de les accompagner avec efficacité dans leurs projets et de les préparer convenablement au monde de la défense nationale. C'est pourquoi il serait préférable d'envisager une période de six mois, tout en tenant compte des problématiques liées au calendrier universitaire, à la signature de contrats de travail ou d'alternance. Surtout, faire dans la demi-mesure coûterait cher pour peu de résultats. Si nous voulons donner à ces jeunes les moyens de réussir, alors allons jusqu'au bout, avec un budget adéquat. Certes, les contraintes budgétaires sont réelles, mais il s'agit avant tout d'un effort pour la Nation, un choix d'avenir. Enfin, je tiens à le souligner, il existe des dispositifs qui fonctionnent très bien dans notre pays. Je pense aux centres du service militaire volontaire, en particulier celui de Brétigny-sur-Orge, qui opèrent un travail remarquable au niveau de l'insertion professionnelle et offrent ainsi une seconde chance à ces filles et ces garçons. Il pourrait donc être intéressant, une fois les objectifs déterminés, de s'orienter vers ce type de mesure, où l'association du militaire et du civil fonctionne parfaitement, où la mixité est rendue possible au travers, notamment, d'échanges avec des élèves issus de grandes écoles.

Comme vous l'indiquez dans votre question, le Président de la République s'est engagé à renforcer le lien entre l'armée et la jeunesse et, plus largement, à développer le sentiment d'appartenance à la Nation de notre jeunesse par la création d'un service national universel, service national universel, qui sera marqué du sceau de l'engagement. Aussi, le Premier ministre a nommé en septembre dernier une mission interministérielle composée des inspections générales des ministères concernés pour dresser un état des lieux des nombreux dispositifs existants- ils sont très nombreux -, les évaluer et formuler des propositions. Le rapport a été remis au début du mois de novembre. D'autres travaux menés parallèlement par les députés et les sénateurs vont permettre d'enrichir la réflexion du Gouvernement. À ce stade, certains présupposés paraissent incontournables : le dispositif aura vocation à contribuer à la résilience de la Nation et à permettre un brassage social de la jeunesse il revêtira un caractère interministériel au regard des nombreuses contributions dont il bénéficiera ; il permettra de développer l'esprit de défense, de valoriser les métiers des armées et d'en renforcer l'attractivité il s'agira d'un dispositif en adéquation avec les objectifs et les moyens de l'État ; l'engagement des jeunes au profit de la société sera valorisé. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un projet de société d'envergure- on compte, je le rappelle, 800 000 jeunes par tranche d'âge -, qui nécessite du temps et une concertation avec tous les acteurs directement intéressés.

Enfin, comme vous, le Gouvernement est mobilisé pour l'insertion professionnelle des jeunes. C'est pourquoi le dispositif du service militaire volontaire

rappelle que le démantèlement des campements près de Calais et le renfort des effectifs pour sécuriser les accès au tunnel sous la Manche n'ont pas pour autant fait disparaître les migrants, les conduisant à se déplacer. Dans le Calvados, des communes littorales comme Ouistreham, petite ville portuaire, voient arriver de plus en plus de clandestins candidats au départ pour l'Angleterre- surtout depuis le démantèlement de la « jungle » calaisienne et le rétablissement des contrôles aux frontières. Il s'agit de jeunes hommes, parfois mineurs, originaires du Soudan ou d'Érythrée, désireux de s'embarquer par tout moyen sur les navires de la liaison maritime entre Ouistreham et Portsmouth assurée par la compagnie Brittany Ferries. Des groupes d'individus, démunis, sont régulièrement signalés, errant en ville ou cachés sur des chantiers, dans des jardins ou sous des haies. Ils survivent dans des conditions précaires, en particulier durant la période hivernale. Ce flux de migrants, en augmentation croissante ces derniers mois, crée tensions et inquiétudes auprès de la population. La situation n'est satisfaisante sur le plan ni humanitaire ni sécuritaire. Quant à l'économie locale, elle se détériore par la baisse des ventes dans les commerces de la ville. De plus, des ventes de commerces et de biens immobiliers ainsi que des réservations d'hébergements touristiques sont annulées. Ouistreham, beaucoup ont en mémoire la détresse des habitants de Calais face au marasme de leur ville et craignent une crise migratoire qui s'installe dans la durée. Il est impératif de mettre un terme à cet odieux trafic d'êtres humains sur notre territoire et de ne pas laisser se créer de nouveaux points de fixation. Madame la secrétaire d'État, quels sont les résultats concrets obtenus à l'encontre des réseaux de traite des êtres humains opérant dans ou vers le Calvados ? Quelles mesures supplémentaires le Gouvernement entend-il prendre pour lutter

d'État auprès de la ministre des armées. Monsieur Allizard, les routes et les modes opératoires utilisés par les migrants souhaitant se rendre illégalement au Royaume-Uni, souvent guidés par des réseaux de passeurs sans scrupule, vous l'avez dit, varient. En conséquence, les autorités françaises adaptent leurs réponses afin de lutter contre les filières d'immigration irrégulière, de prévenir les franchissements illicites de la frontière et de garantir l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. Afin de contrecarrer l'activité des réseaux de passeurs, un travail impliquant l'ensemble des services de police et de gendarmerie est mené avec l'institution judiciaire. Dans l'ensemble de la zone de défense « ouest », quinze filières ont ainsi été démantelées de janvier à septembre 2017, soit une progression de plus de 36 % par rapport à la même période en 2016. La pression migratoire constatée dans le Calvados, et plus particulièrement au port de Ouistreham, s'est en effet accrue au cours des dernières semaines. L'action des forces de sécurité intérieure a été orientée en conséquence : trente-huit militaires du groupement de gendarmerie du Calvados interviennent quotidiennement pour empêcher les tentatives d'intrusion dans l'emprise du port et contrôler la régularité du droit au séjour des personnes interpellées, avec le renfort de seize réservistes opérationnels, de seize gendarmes mobiles et le soutien d'un demi-escadron de gendarmes mobiles qui sera maintenu tant que cela sera nécessaire. Les militaires de l'opération Sentinelle interviennent également en soutien. Enfin, il importe de dissuader les tentatives de franchissement illégal de la frontière franco-britannique par une sécurisation accrue des emprises portuaires. À cette fin, le Gouvernement a sollicité et obtenu du gouvernement britannique une contribution financière au renforcement des infrastructures de plusieurs ports de la Manche. Dans ce cadre, 2,44 d'euros sont alloués à la sécurisation du port de Ouistreham, notamment pour l'acquisition de systèmes de détection, la création d'un hangar d'inspection filtrage ainsi que l'installation de clôtures, de portails et de systèmes de vidéosurveillance. Ces travaux de sécurisation seront engagés au cours des prochaines semaines. La parole

du nettoyage ou de l'accroissement des patrouilles de police municipale. Rien que pour une petite ville comme Ouistreham, le coût supplémentaire s'élevait à 100 000 euros pour 2017, à un moment où les dotations de l'État aux collectivités diminuent. Par ailleurs, et vous l'avez souligné, les stratégies des réseaux de passeurs sont de plus en plus élaborées, ce qui rend les opérations de police d'autant plus compliquées. Ce qui nous inquiète également, c'est que des trafics s'organisent désormais sur nos aires d'autoroutes la nuit, mettant en péril la sécurité tant, certes, des migrants que des usagers ; c'est un fait avéré. un fait avéré. Des migrants ont déjà été condamnés en correctionnelle à Caen pour des violences sur les forces de l'ordre. La situation déborde d'ailleurs largement sur Caen et sa proche périphérie, où se créent des points de regroupement de migrants dans lesquels les trafics et la misère prospèrent. Nous souhaiterions que l'État en prenne toute la mesure. La seule augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, que je salue par ailleurs- elle était nécessaire -, ne pourra pas tout résoudre. Au-delà de la France, c'est bien, je le crois, l'Union européenne qui est face à une crise migratoire qu'elle a laissé s'amplifier. Une plus grande fermeté et un meilleur respect des règles d'entrée et de séjour dans l'Union européenne, ainsi

dans la prise en charge des migrants. Je souhaite que le sommet franco-britannique prévu jeudi traite également de ce sujet. Je crois que nous n'échapperons pas à une réflexion sur la remise en cause ou, en tout cas, sur la renégociation des accords du Touquet. Nous en